est une technique qui consiste, pour un commercial, à solliciter par téléphone quelqu’un qui n’a pas manifesté d’intérêt pour les produits ou services qu’il vend. de loi vise à mettre fin au démarchage téléphonique tel qu’il vient d’être défini. Je sais, madame la rapporteure, que la définition du n’est pas la même que celle du droit commercial ou du droit de la concurrence. Ce sujet soulève une question qui traverse toutes les sociétés modernes : celle de la gestion de nos données personnelles, qui sont captées, légalement ou non, vendues, échangées, utilisées, stockées.

et un téléconseiller, souvent installé de l’autre côté de la Méditerranée, essaie alors d’engager la conversation afin de nous vendre quelque chose. Quelle est la situation ?

ce qui signifie que chaque Français est considéré comme consentant au démarchage téléphonique. Depuis un certain nombre d’années, des lois ont été votées, des décisions ont été prises, afin d’essayer de réguler, d’encadrer et de contraindre les acteurs du marché.

La vérité, c’est que le démarchage téléphonique à froid ne fonctionne plus. Comme dirait le dicton populaire : trop de démarchage tue le démarchage. J’en veux pour preuve ce que beaucoup d’entreprises sérieuses nous ont dit au cours de nos travaux

pourtant rien demandé, ne comprennent pas comment leur numéro a pu être communiqué et sont impuissants à faire respecter leur tranquillité. Ils en ont marre, et nous sommes quelques uns dans cet hémicycle à partager ce sentiment. Selon UFC Que Choisir, 97 % des Français sont exaspérés par le démarchage téléphonique. Les associations de consommateurs que j’ai auditionnées ont unanimement confirmé que ledit démarchage faisait partie de ces irritants du quotidien qui nous empoisonnent la vie. C’est dans ce contexte que notre collègue Pierre Jean Verzelen a déposé une proposition de loi visant à interdire cette pratique, du moins à en resserrer drastiquement l’encadrement. Cette volonté de s’attaquer une nouvelle fois au fléau du démarchage téléphonique abusif doit être saluée,

Le démarchage téléphonique légal, mais non sollicité, doit être distingué de deux phénomènes connexes, qui lui sont pourtant largement associés dans l’esprit des consommateurs en raison de la similarité des nuisances qu’ils engendrent. tout d’abord du démarchage électronique, par mail ou par SMS, qui est soumis à un régime juridique distinct et qui repose sur le principe de l’. La légalité de l’opération est alors conditionnée au consentement

Ce cadre législatif a été significativement renforcé en 2020, notamment grâce à l’apport de notre collègue André Reichardt. Hélas, la loi Naegelen n’a pas produit les résultats que nous espérions

les sanctions sont insuffisantes. Certes, 200 amendes administratives ont été prononcées l’année dernière pour un montant total de 4,4 millions d’euros, mais les mailles du filet sont larges… Sur ce point, ne nous leurrons pas : la persistance des nuisances résulte moins d’éventuelles lacunes du cadre juridique que d’une masse de comportements voyous de la part d’acteurs souvent situés à l’étranger et parfaitement indifférents à leurs obligations légales. que le déploiement des solutions techniques prescrites par le législateur pour limiter les nuisances est totalement embourbé. La loi Naegelen imposait aux opérateurs de déployer un mécanisme d’authentification

bref, nous sommes soumis au bon vouloir d’opérateurs, qui ont eux mêmes abondamment recours au démarchage. Je me permets d’attirer votre attention, madame la secrétaire d’État, sur cette situation profondément regrettable.

Alors que cette ultime tentative de sauvetage de l’ a échoué, l’ est désormais la seule solution qui nous reste. Nous devons prendre acte de l’épuisement de l’ensemble des autres options disponibles pour répondre à l’exaspération légitime de nos compatriotes.

Pour surmonter ces obstacles, je vous soumettrai un amendement visant à aligner le régime du démarchage téléphonique sur celui du démarchage électronique. De la sorte, la lisibilité du cadre juridique d’ensemble sera renforcée, tandis que les effets sur l’emploi seront maîtrisés.

propose ainsi, d’une part, de réduire la fréquence et les horaires d’appel autorisés, de l’autre, d’interdire explicitement le rappel d’un consommateur ayant exprimé son refus d’être démarché au cours de la conversation. Deuxièmement, il faut protéger les consommateurs les plus vulnérables. Les personnes âgées sont bien souvent les premières victimes de démarcheurs « cow boys » peu scrupuleux. Pour les protéger, je propose d’introduire un délai de carence de vingt quatre heures avant l’acceptation d’une offre commerciale transmise par téléphone. Je propose également de renforcer les sanctions pour les faits d’abus de faiblesse lorsqu’ils sont commis par l’entremise d’un démarchage téléphonique. Troisièmement, il convient de mieux maîtriser l’utilisation des données des consommateurs. Je propose que leur consentement soit requis pour l’inscription de leur ligne fixe dans l’annuaire, comme c’est le cas pour les mobiles. souhaite faciliter la tâche des administrations pour poursuivre et sanctionner. Toutes m’ont alertée sur les difficultés qu’elles rencontraient à se partager des informations pourtant cruciales, en raison du secret de l’instruction. Je proposerai en outre de modifier le titre de la proposition de loi pour éviter tout risque de déception des consommateurs. Vous l’aurez compris, la commission des lois est pleinement associée à la démarche de notre collègue Pierre Jean Verzelen dans la lutte contre les nuisances associées au démarchage téléphonique abusif. La parole

Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous serons tous d’accord pour dire que le démarchage téléphonique préoccupe un nombre important de Français. Il constitue aujourd’hui un irritant de la vie quotidienne sur lequel nous sommes, les uns et les autres, régulièrement interpellés.

le maire d’une commune rurale me disait récemment qu’il n’arrivait plus à joindre certains de ses concitoyens en cas de difficultés particulières, par exemple météorologiques, parce que certaines personnes âgées ne décrochent plus leur téléphone du fait de ce harcèlement. Je remercie donc le sénateur Verzelen de mettre ce sujet à l’ordre du jour. Je voudrais commencer par rappeler quelques points importants. Le démarchage téléphonique en France est légal et autorisé ; par exception, il est interdit dans certains cas de figure,

l’ensemble des Français qui ne souhaitent plus être démarchés à s’y inscrire. Le dispositif commence à être connu, mais il peut encore gagner en notoriété.

Premièrement, la prospection téléphonique a été interdite pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Cette interdiction a ensuite été étendue aux appels relatifs au compte personnel de formation.

Troisièmement, la loi a prévu des sanctions plus dissuasives en cas de manquement. Elle retient désormais la responsabilité du donneur d’ordre des appels émis.

: s’ils constatent que le numéro ne correspond pas à l’identité de celui à qui il a été attribué, c’est à dire qu’il y a usurpation, ils doivent bloquer l’appel.

Des contrôles de la DGCCRF sont activement menés ; j’en profite pour rappeler à nos concitoyens qu’ils peuvent signaler, soit sur Bloctel, soit sur SignalConso, les appels frauduleux qu’ils reçoivent.

demande. Malgré cela, force est de constater que de nombreuses pratiques illégales perdurent. Je crois que nous devons d’abord mieux les connaître et les identifier pour pouvoir agir efficacement.

le délai a donc été prolongé jusqu’au 1 octobre 2024. Depuis cette date, vous avez suivi dans la presse un certain nombre d’évolutions : il semble que les opérateurs parviennent à bloquer les appels usurpés lorsqu’ils sont à destination d’un téléphone fixe. C’est une première avancée. Pour autant, le mécanisme ne fonctionne pas lorsque l’appel se dirige vers un téléphone mobile. C’est bien évidemment un sujet de préoccupation essentielle compte tenu de l’équipement en téléphones mobiles de nos concitoyens…

c’est que les fraudeurs contre lesquels nous souhaitons tous lutter – et je rappelle que les services de l’État et de la DGCCRF sont fortement mobilisés

Deuxième difficulté, la proposition de loi présente un certain nombre de fragilités juridiques. Elle interdit rigoureusement tout démarchage téléphonique, y compris celui qui est effectué dans de bonnes conditions

du mécanisme d’authentification des numéros. La loi a été votée en 2020 ; quatre ans plus tard, le déploiement est partiellement engagé, mais chacun mesure les progrès qui restent à faire.

en juillet dernier, dans le Nord, un retraité a été dépouillé de 70 000 euros après avoir été victime d’une escroquerie bien orchestrée : d’abord démarché par téléphone, il a ensuite remis sa carte bancaire à un faux coursier, qui a vidé ses comptes sans scrupules. Ce fait divers n’est malheureusement qu’un exemple parmi tant d’autres des dérives que le démarchage téléphonique peut engendrer. Ce dernier est juridiquement défini à l’article L. 221 16 du code de la consommation comme le fait pour un professionnel de contacter un consommateur en vue de conclure un contrat. Selon une récente enquête de l’UFC Que Choisir, 92 % des Français se disent dérangés par les nuisances du démarchage téléphonique, ce qui illustre le fait que la réglementation en vigueur ne suffit manifestement pas à protéger efficacement les consommateurs. Depuis une dizaine d’années,

Ainsi, la loi Hamon de 2014 a introduit un droit d’opposition dans le code de la consommation. Depuis, l’inscription sur la liste Bloctel est censée permettre de ne plus recevoir d’appels non sollicités. Dans les faits, seulement 2 400 entreprises, 6 millions de consommateurs et 12 millions de numéros de téléphone y sont répertoriés en 2024, ce qui ne représente que 9 % des Français et 10 % des lignes téléphoniques. Après la loi Hamon, un autre texte, issu de la

et de la distribution de la presse) et la Cnil sont régulièrement sollicitées pour des plaintes et signalements pour démarchage abusif. Et les sanctions prévues, bien qu’élevées, ne sont que rarement appliquées, faute de contrôles adaptés.

tel régime s’applique déjà en matière de rénovation énergétique ou de compte personnel de formation, pour lesquels tout démarchage est interdit sans consentement. En Allemagne, tout démarchage téléphonique sans consentement préalable est illégal et les entreprises contrevenantes risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 euros.

pourraient eux aussi exprimer explicitement leur consentement avant d’être démarchés téléphoniquement. C’est une position que les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain défendent avec constance et qu’ils ont rappelée en 2020, lors des débats sur la proposition de loi Naegelen. Cette position semble désormais incontournable face à l’épuisement des autres options, comme l’a également souligné la rapporteure Olivia Richard. Bien évidemment, ce consentement préalable doit lui même être exprimé dans le respect des règles de protection des données personnelles et de liberté d’information, de consommation comme d’entreprendre. Aussi, nous souscrivons aux propositions de réécriture du texte dont l’idée initiale – l’inscription sur une liste – n’apparaît pas robuste juridiquement. Les amendements de la rapporteure visant à aligner le consentement au démarchage téléphonique sur le consentement au démarchage électronique nous paraissent pertinents,

en encadrant mieux le démarchage téléphonique « officiel », comme nous entendons le faire ce matin, nous ne ferons pas disparaître d’un coup tout démarchage frauduleux – j’ai d’ailleurs déposé un sous amendement sur cette question. Les appels sur les lignes fixes et mobiles ne cesseront pas totalement pour qui n’a pas donné son consentement préalable, mais au moins l’on saura que, sauf presse, association ou relation contractuelle préexistante, ils sont forcément le fait de fraudeurs. On pourra donc plus facilement les dénoncer. À cet égard, il est possible de rassurer les représentants des territoires et des entreprises qui craindraient l’effet négatif sur l’emploi de l’adoption de la présente

Nous pensons donc sincèrement, madame la secrétaire d’État, que nous pouvons préserver nos emplois tout en protégeant mieux les consommateurs, notamment ceux qui sont constamment dérangés, que ce soit sur leur téléphone fixe ou sur leur portable. C’est en ce sens que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutient les dispositions qui permettront, demain, de passer à un démarchage téléphonique consenti pour tous et de soulager le quotidien de nos concitoyens, exaspérés par ces dérangements intempestifs

de nombre de nos concitoyens, le législateur a tenté, depuis plusieurs années, d’encadrer chaque fois un peu plus cette pratique.

Dès 2016, un dispositif gratuit d’opposition au démarchage téléphonique – Bloctel – a été mis en service. Toutefois, force est de constater que seuls 9 % des Français sont inscrits sur cette plateforme en 2024 et que les appels intempestifs continuent de plus belle… 2020, deuxième tentative : Bloctel n’ayant pas résolu le problème, la loi du 24 juillet renforce l’encadrement du démarchage, qui est désormais interdit dans le secteur de la rénovation énergétique et de la formation. Mais, de nouveau, cela ne suffit pas. Alors, en 2023, un décret est venu préciser les plages horaires et les jours pendant lesquels le démarchage est autorisé. Ce décret fixe aussi des règles relatives aux fréquences des appels.

Sans changement de paradigme, nous ne pouvons espérer que les Français ne soient plus sursollicités, voire harcelés. C’est tout le sens de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Plutôt que d’autoriser le démarchage en y apportant, à chaque fois, un peu plus de limites, ce texte propose d’inverser le principe en interdisant le démarchage, quelques exceptions.

Par principe, tout démarchage téléphonique est qualifié de harcèlement inacceptable et interdit auprès de tout consommateur qui n’y aurait pas donné son consentement explicite préalable. L’article unique de cette proposition de loi vise également à interdire le démarchage téléphonique, à l’exception de trois cas : si la personne s’est inscrite sur une liste de consentement ; dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours

C’est parce que le démarchage empoisonne la vie des Français, qui ne font plus la distinction entre démarchage régulier et démarchage intempestif ou frauduleux,

Pour beaucoup, c’est une gêne ; pour d’autres, en particulier les personnes âgées et vulnérables, c’est une source d’exaspération. Pourtant, voilà plusieurs années que les pouvoirs publics et le législateur tentent de réguler cette pratique et de mettre un terme à une à une telle dérive commerciale. Certes, chaque consommateur peut référencer son numéro sur une liste pour éviter les appels intempestifs. Toutefois, depuis 2016, le fameux dispositif Bloctel, qui devait permettre aux consommateurs inscrits volontairement de s’opposer au démarchage téléphonique, a largement fait les preuves de ses limites. Et même s’il donne quelques résultats, beaucoup de particuliers ne connaissent toujours pas son existence ou son fonctionnement. J’ajoute que nombre d’entreprises de vente directe s’affranchissent, souvent délibérément, de consulter la liste des numéros inscrits sur Bloctel avant de démarcher un éventuel client. À l’été 2020, le Parlement avait pourtant adopté une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Malgré cela, la DGCCRF, en intensifiant ses contrôles, a relevé plusieurs milliers d’infractions. Certes, des sanctions ont été prises à la suite de certaines enquêtes. Par exemple, en août dernier, une société de conseil s’est vu infliger une amende administrative de 300 000 euros pour, notamment, ne pas avoir respecté l’interdiction de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. De manière générale, les infractions constatées sont principalement liées au non respect de l’inscription sur Bloctel, à des démarchages dans des secteurs proscrits ou durant des périodes non autorisées par le décret du 13 octobre 2022, qui interdit toute prospection commerciale le week end

72 % des Français se disaient démarchés au moins une fois par semaine sur leur téléphone portable et – encore plus inacceptable ! – 38 % au quotidien. En moyenne, chaque Français reçoit environ six appels de démarchage par semaine. Les secteurs les plus cités sont l’assurance, les placements financiers et la rénovation énergétique – le démarchage dans

En adoptant la loi du 24 juillet 2020, le législateur n’avait finalement pas osé remettre en cause le régime d’opposition expresse, dit, considérant à l’époque que le consentement préalable du consommateur – – reviendrait à faire disparaître le secteur économique du démarchage et ses emplois. Je crois indispensable aujourd’hui de prendre acte de l’inefficacité de la logique du droit d’opposition. Fort de ce constat d’échec, il faut opérer un changement en posant désormais le principe d’un explicite, dans lequel chaque consommateur doit donner individuellement son consentement préalable pour être contacté par téléphone,

En Allemagne, par exemple, ce consentement, qui ne peut être ni implicite ni déduit d’une relation existante, revêt plusieurs formes : un formulaire en ligne ou papier ; une inscription sur un site ou à un service ; un accord explicite lors de contrats commerciaux. Ces contraintes n’ont pas entraîné de séisme économique dans le secteur du marketing à distance. Les entreprises concernées interagissent avec les consommateurs qui en ont fait le choix le choix et continuent d’assurer le suivi de leurs relations commerciales. Rien ne s’oppose donc véritablement à ce principe clair : aucun consommateur ne doit être contacté par une entreprise de démarchage téléphonique sans l’avoir explicitement consenti.

que si les sanctions prévues pour les professionnels ne respectant pas ces règles sont suffisamment dissuasives et réellement appliquées. Cette proposition de loi prévoit des montants d’amende élevés ; cela implique que la DGCCRF dispose de moyens significatifs pour mener de multiples contrôles et traiter les plaintes. C’est sur ce point qu’il nous faudra être particulièrement vigilants. Resterait probablement une question : une part non négligeable du démarchage illicite provient de centres d’appels situés à l’étranger. Ils échappent ainsi plus facilement à la réglementation française, aux contrôles et donc aux sanctions. Il convient enfin de rappeler que, au delà du démarchage abusif, les entreprises de vente directe ont aussi l’obligation de respecter certaines règles commerciales, comme la bonne information du consommateur sur leur droit de rétractation.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi qui vise à répondre à un fléau que nous connaissons tous trop trop bien : le démarchage téléphonique intempestif. Ce phénomène touche des millions de nos concitoyens et suscite une exaspération légitime. Près de 72 % des Français sont démarchés au moins une fois par semaine sur leur portable et 38 % subissent ces appels quotidiennement. La situation est tout aussi préoccupante pour les lignes fixes, où le taux de démarchage hebdomadaire atteint 58 %. La loi Hamon de 2014 a mis en place un régime d’, permettant permettant aux consommateurs de s’inscrire sur la liste Bloctel pour s’opposer au démarchage. Cependant, malgré plus de 12 millions de numéros recueillis, ce dispositif ne couvre que 10 % des lignes téléphoniques. Par ailleurs, les signalements à la DGCCRF montrent que de nombreux professionnels, notamment ceux qui opèrent depuis l’étranger, contournent ces règles. La loi Naegelen de 2020 a cherché à renforcer ce dispositif en encadrant les horaires et la fréquence des appels. Les sanctions ont été durcies, mais restent encore trop faibles pour être dissuasives : en 2023, seulement 200 amendes ont été prononcées pour un total de 4,4 millions d’euros, ce qui est bien

où chacun doit s’inscrire pour bloquer les appels, à un régime d’, interdisant par principe le démarchage sans consentement préalable. Ce modèle, déjà en vigueur pour la prospection électronique, permettrait de faire respecter un droit fondamental des consommateurs : celui de contrôler leur tranquillité et leur vie privée. Le texte prévoit également des exceptions pour les clients existants, pour les associations, pour les sondages et pour la presse, tous secteurs pouvant justifier des contacts avec les consommateurs. Cependant, des objections ont été soulevées lors de l’examen en commission, notamment quant à la faisabilité juridique et aux répercussions économiques de ce changement. Le RGPD impose un consentement spécifique, ce qui rend difficile la mise en place d’une liste de consentement universelle. De plus, cette transition pourrait affecter les quelque 29 000 à 40 000 emplois du secteur, même si les acteurs concernés estiment qu’une adaptation des pratiques permettrait de sauvegarder l’emploi.

au cas par cas par chaque entreprise, serait davantage compatible avec le RGPD et préserverait des emplois en laissant les entreprises adapter leurs méthodes de contact. Cet amendement tend également à prévoir une entrée en vigueur au 11 août 2026 coïncider avec la fin de la concession actuelle de Bloctel, ce qui assurera une transition progressive pour les opérateurs. Si les ajustements proposés sont intégrés au texte, notre groupe soutiendra cette évolution législative, qui répond à une attente forte. Nous espérons que ce cadre permettra de protéger les citoyens contre des pratiques envahissantes, tout en préservant les acteurs économiques respectueux de la loi. Nous sommes convaincus qu’avec ces modifications nous pourrons avancer vers un modèle qui protège efficacement la vie privée des consommateurs, tout en assurant la viabilité des entreprises de démarchage responsables. La parole

mes chers collègues, le constat est simple : la grande majorité des Français ne répondent plus au téléphone quand un numéro inconnu les appelle. Quelque 500 000 personnes sont victimes d’arnaques téléphoniques chaque année. Certains de nos concitoyens sont confrontés quotidiennement à des démarchages abusifs. Autant dire que cette proposition de loi a le grand mérite de mettre sur la table une problématique du quotidien. Le dispositif Bloctel, issu de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, a permis au consommateur de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels

Jusqu’à présent, toutes les évolutions législatives se sont construites autour d’un principe commun : elles présument du consentement du consommateur à être démarché, puisque c’est à lui qu’il revient d’exercer son droit d’opposition au démarchage. Seulement, les abus que nous constatons nous imposent de changer de braquet. Et ce changement devra être législatif, mais pas exclusivement. Il faudra se donner les moyens de l’appliquer efficacement et avec dureté à l’égard des entrepreneurs peu scrupuleux. Évidemment, il y a un sujet économique et social. Le démarchage téléphonique représente des emplois ; il constitue même un outil clé dans certains secteurs d’activité. Le législateur ne l’a jamais ignoré, puisque toutes les mesures de lutte contre le démarchage abusif ont reconnu certaines exceptions : les appels des professionnels avec lesquels les consommateurs ont des relations contractuelles préexistantes les appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines ; ou encore les appels émanant d’instituts d’études et de sondages, d’associations à but non lucratif ou d’un service public. Or, en l’état actuel des choses, ces exceptions se retrouvent noyées dans la masse des appels. Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre une politique publique efficace pour protéger autant le consommateur que les entreprises qui vivent d’une forme saine de démarchage. Le texte initial présenté par notre collègue Pierre Jean Verzelen avait peut être des défauts rédactionnels, mais il présentait la grande qualité de poser le problème dans des termes clairs et explicites. Aussi, je veux saluer le travail de notre rapporteure Olivia Richard et de la commission des lois qui permet de poursuivre l’initiative et de mieux mettre en musique ces propositions.

mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue Pierre Jean Verzelen concerne une réalité qui incommode chaque jour nos concitoyens. Je le remercie pour cette initiative, car le démarchage téléphonique est une préoccupation réelle et, bien souvent, une cause d’exaspération largement partagée. Porté par une volumétrie massive, le démarchage téléphonique peut en outre constituer une menace pour les publics fragiles et relayer des arnaques.

Le développement des moyens de communication est évidemment un vecteur de développement économique. Cependant, l’alliage du démarchage téléphonique, d’une part, et de la prospection commerciale à forte intensité, de l’autre, ne présente pas que des avantages. Je dirai même plus : nos concitoyens disent stop Réalité ancienne, le démarchage téléphonique à finalité commerciale s’est fortement développé ces vingt dernières années. Il est tous azimuts – ou presque –, il met en péril la tranquillité de nos concitoyens, il sature leurs flux téléphoniques et il met en situation de vulnérabilité les publics les plus fragiles. Les données personnelles sont devenues autant de renseignements marchands brassés par les opérateurs sans que les détenteurs de téléphones, qu’ils soient fixes ou mobiles, aient donné un quelconque accord. Nous sommes tous contactés, parfois plusieurs fois dans la journée, par des numéros tantôt masqués, tantôt inconnus, pour différents services ou prestations. Ces appels répétitifs sont gênants. Ils présentent un caractère intrusif. Ils peuvent en outre constituer un piège : les associations de défense des consommateurs et des usagers sont unanimes sur ce sujet et interpellent régulièrement les pouvoirs publics. De plus en plus de personnes refusent désormais de décrocher, redoutant un énième appel de démarchage. Nous pouvons donc l’affirmer, ce phénomène constitue, à bien des égards, une source de nuisances. Des mécanismes législatifs ont pourtant été introduits pour réguler et encadrer le démarchage téléphonique. Cependant, force est de constater qu’ils sont très largement inefficaces. La liste d’opposition Bloctel demeure ainsi confidentielle et limitée. Quelles que soient les démarches des consommateurs, elle est malheureusement, dans les faits, peu efficace. Madame

Ce cadre est à la fois plus respectueux de la vie privée et constitue un bouclier efficace. Ce qui nous rassemble sur cette proposition de loi, c’est la recherche du juste équilibre entre la vie économique et le domaine des télécoms, d’un côté, et la prévention des sollicitations intempestives de l’autre. Nous devons gagner en efficacité à cet égard. La proposition de loi de notre collègue vise à instaurer un changement de perspective. Les motifs qui poussent à changer de braquet sont à nos yeux fondés. Il s’agit de passer d’une logique générale d’acceptation tacite du démarchage par le consommateur avec possibilité d’opposition, à une logique générale d’opposition avec possibilité de consentement explicite. La préservation de l’emploi et la stimulation du tissu économique sont des objectifs partagés par tout le monde dans cet hémicycle. Comme cela a été souligné et documenté en commission, la plupart des appels sont cependant passés depuis des centrales à l’étranger,

dans le cadre des exceptions que le texte prévoit lui même puisqu’ils concernent des relations commerciales approfondies. Mes chers collègues, les mécanismes proposés dans la proposition de loi sont restrictifs et entraîneront sans doute certaines recompositions pour ces organismes de démarchage. Ils disposeront d’autres relais,

Ces propositions ont été discutées au sein de la commission des lois. Un consensus semble émerger pour soutenir ce texte, en constante amélioration depuis qu’il a été déposé, en particulier pour définir collégialement des modalités pratiques de recueil du consentement des usagers et des consommateurs, en conformité avec le RGPD. Aujourd’hui, le groupe Union Centriste estime que les tentatives d’encadrement et de régulation n’ont pas produit les résultats escomptés et que la lassitude de nos concitoyens doit être pleinement prise en compte. Nous devons notamment mieux protéger

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que plusieurs lois et décrets ont tenté, par le passé, d’encadrer le démarchage téléphonique, nous partageons aujourd’hui le même constat ces mécanismes n’ont pas limité cette pratique et ses conséquences. Neuf Français sur dix sont toujours exaspérés par le démarchage téléphonique. Et pour cause : 72 % des Français sont démarchés au moins une fois par semaine, 38 % quotidiennement.

alors que 97 % des Français sont exaspérés par les démarchages téléphoniques, seulement six millions de nos concitoyens sont inscrits sur Bloctel. Si l’on peut s’interroger sur le manque de communication sur ce dispositif, c’est surtout son efficacité qui semble faire défaut.

Et les sanctions sont insuffisantes au regard des millions d’appels passés. Pourtant, le démarchage téléphonique n’est pas qu’exaspérant ; il est aussi dangereux, particulièrement pour les plus vulnérables. Les centres d’appels le reconnaissent eux mêmes : ils visent essentiellement les personnes fracturées électroniquement. Or c’est 18 % de la population française qui est en situation d’illectronisme, les personnes âgées étant Combien parmi nous ont un parent ou un ami ayant été victime d’une arnaque téléphonique ? En Europe, en 2023, 16 % des consommateurs

L’UFC Que Choisir le demande déjà depuis plusieurs années, au nom du droit à la tranquillité. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait une dizaine de pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche, la Lituanie ou la République tchèque. Il nous faut inverser la pratique et ne plus faire peser sur les consommateurs la charge de se prémunir contre le démarchage. C’est bien le rôle du droit que de protéger les personnes les plus vulnérables. Avec l’interdiction par défaut des démarchages téléphoniques, les entreprises ne pourront contacter que des personnes inscrites sur une liste et ayant, pour parler en termes contractuels, consenti à la démarche. Cela permettra de fortement réduire ce qui exaspère, je le répète, 97 % de nos l’avenir, si vous faites l’objet d’un démarchage téléphonique, mais que vous n’êtes pas inscrit sur la liste, vous saurez que la démarche est illégale. Mes chers collègues, si les entreprises ont des droits, les citoyens en ont aussi. Est on un consommateur avant d’être un citoyen ? Je ne le pense pas.

tous les orateurs qui m’ont précédée – c’est le problème de passer en dernier –, le démarchage téléphonique est incontestablement une nuisance. Les appels non sollicités viennent interrompre des tâches quotidiennes, dérangent lors d’un dîner ou pendant les congés.

décrets. Pourtant, nous sommes toutes et tous toujours démarchés. Pourquoi ? Est ce parce qu’il serait impossible d’interdire le démarchage téléphonique ? Non, un seul article de loi suffit. D’ailleurs, de nombreux pays européens, comme le Portugal et l’Allemagne, l’ont interdit depuis longtemps.

l’ont fait. Je ne vais pas balayer cet argument d’un revers de main ; je vais plutôt essayer de l’analyser. Le problème, c’est que cette analyse, qui devrait comprendre une étude des conditions de travail des opératrices et des opérateurs téléphoniques n’est pas souvent fournie par celles et ceux qui avancent cet argument. Quand on s’intéresse à cette question, on ne peut que constater que ces opérateurs, quand ils bénéficient du statut de salarié, sont extrêmement mal payés, subissent une pression énorme de leur hiérarchie, souffrent du manque de sens de leur activité et d’un mal être au travail qui les conduit bien souvent à la dépression.

et la nécessité de faire évoluer le système existant. Je pense que tout le monde en convient. À cet égard, je tiens à saluer l’initiative de l’auteur de la proposition de loi, ainsi que le travail de notre rapporteure, Olivier Richard. Cet amendement a été élaboré par mon collègue André Reichardt,

Par ailleurs, nous nous appuyons sur un dispositif juridique solide en matière de consentement en nous rapprochant de celui du RGPD, lequel exige un consentement non pas général, mais bien spécifique.

puisqu’ils nous permettent de trouver des modalités opérantes pour passer du droit d’opposition au consentement préalable. Par ce sous amendement, notre groupe propose simplement deux clarifications. La première porte sur le RGPD. Il nous semble que nous ne sommes pas

des numéros. À cet effet, nous rassemblerons prochainement tous les opérateurs téléphoniques pour faire un point d’étape sur ce sujet. Pour autant, ces deux amendements nous semblent ouvrir une perspective utile. Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse.

de petits malins pourraient faire du consentement au démarchage téléphonique une condition préalable à l’achat de leurs produits et l’introduire dans leurs conditions générales de vente. C’est pour éviter cela et pour que l’article que nous venons d’adopter soit pleinement efficace que nous proposons de compléter la liste des pratiques commerciales interdites. Il serait ainsi interdit, conformément à la volonté que nous venons d’exprimer, de conditionner l’achat d’un bien ou d’un service au consentement au démarchage téléphonique.

du RGPD. La Cnil précise bien qu’une « personne doit se voir offrir un choix réel sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus ». Cependant, le passage à l’va engendrer un bouleversement important. Il n’est donc pas inutile de faire œuvre de clarté sur ce sujet, comme l’a souligné Mélanie Vogel.

D’abord, le montant des amendes et des peines d’emprisonnement proposées excède largement les quantum prévus dans le code de la consommation. Les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont en effet punies d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

considèrent toutefois que la rédaction figurant actuellement dans le code de la consommation est trop restrictive pour étendre ces dispositifs de filtrage automatisé aux SMS. Il convient donc de lever cet obstacle, étant entendu que les opérateurs demeureront libres de proposer ou non de tels filtres.

C’est une demande très forte de la part de ces instances. En effet, aujourd’hui, le secret de l’instruction fait obstacle à la communication d’informations pourtant cruciales pour le contrôle de la fraude. Ainsi, la DGCCRF ne peut pas signaler à l’Arcep la situation d’un opérateur situé à l’étranger qui utilise un numéro français, en violation du plan national amendement vise également à imposer une obligation de communication à la Cnil des données détenues par les opérateurs, notamment l’identité des affectataires des lignes téléphoniques. La Cnil se voit régulièrement opposer le secret professionnel dans ses enquêtes,

les opérateurs téléphoniques, qui s’appuient sur le diagnostic d’appels automatisés pour les bloquer le cas échéant, ne pourront plus

on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème ». Alors que nous nous apprêtons à examiner le projet de loi de finances pour 2025, je ne crois pas inutile de rappeler cette maxime d’Einstein. Cette année encore, nous voterons un budget en déficit, comme nous le faisons déjà depuis un demi siècle. Cette année encore, nous trouverons en chaque économie un sujet de débat, quand chaque dépense fera l’objet d’un consensus. Cette année encore, nous alerterons sur la dérive de nos finances, mais, au fond, rien ne sera fait pour inverser la donne et engager pour de bon le rétablissement de nos comptes.

Je suis bien marrie de jouer ainsi les Cassandre, mais comment se satisfaire de cette triste pantomime qui, chaque année, se répète et qui, un jour, finira mal ? À mon sens, nous faisons aujourd’hui face à une triple impasse : une impasse financière, une impasse économique et, j’ose le dire, une impasse démocratique. impasse financière, d’abord. Avec une dette publique qui dépasse les 110 % du PIB et un déficit durablement installé au dessus de 5 % du PIB, nous avons renié nos engagements européens, que nous respections encore au début du siècle.

Aujourd’hui, cette réalité déçoit tout le monde. Augmenter les impôts du pays le plus fiscalisé du monde, pour tenir un déficit à 5 % du PIB, tout en rabotant les dispositifs de soutien à l’innovation, c’est mettre notre économie sous forte pression et saper fortement le moral des troupes. Résultat, les investissements et les recrutements sont gelés. La seule chose que les entreprises redoutent plus que les hausses d’impôt, ce sont les hausses d’impôt imprévues,

cette impasse démocratique. Le Parlement pourrait ne plus voter le budget, ce qui est pourtant l’une de ses prérogatives essentielles. En d’autres termes, pour continuer à exercer ses missions, le Parlement devrait en quelque sorte renoncer à exercer son pouvoir. Monsieur le garde des sceaux, vous avez beaucoup œuvré, dans vos précédentes fonctions, au renforcement des mécanismes juridiques, singulièrement organiques, pour améliorer le pilotage de nos finances publiques. Votre rôle aujourd’hui est aussi de veiller au bon fonctionnement de nos institutions. Je me permets donc d’insister sur cette impasse démocratique. En effet, les excellents arguments juridiques que nous entendrons tout à l’heure conduiront de fait à justifier cette situation. Face au constat de cette triple impasse, il serait irresponsable de ne rien faire. Je suis convaincue qu’il est indispensable de changer la méthode par laquelle on élabore le budget.

Le principe en est assez simple. Il s’agit, en matière budgétaire, de donner la primauté à la pluriannualité sur l’annualité. Aujourd’hui, les lois de programmation des finances publiques, prévues par la Constitution, fixent une trajectoire budgétaire que le Gouvernement et le Parlement ont tout loisir, chaque année, de ne pas respecter. Je propose d’inverser la logique, en interdisant l’adoption d’une loi de finances annuelle qui ne respecterait pas la loi de programmation. Cette super loi de programmation pourrait s’intituler « loi portant cadre financier pluriannuel ».

un consensus politique permet tout à fait de s’affranchir de ce cadre. Renforcer la programmation des finances publiques, c’est surtout une mesure de bon sens – et nos concitoyens ont fortement besoin de bon sens. Il s’agit de graver l’engagement au moment où l’ambition est la plus élevée. Le rapporteur général nous le démontre régulièrement : chaque année, les lois de finances s’écartent un peu plus de la trajectoire prévue en loi de programmation. L’adoption d’une telle loi cadre aurait trois principaux effets. Le premier effet serait de contraindre les écarts par rapport à la trajectoire prévue. Le deuxième effet, qui découle du premier, serait de restreindre les débats annuels au périmètre fixé par la loi cadre. Le troisième effet, exigence qui résulte des deux premiers, serait d’améliorer les prévisions macroéconomiques. Ces effets ne sont pas nécessairement souhaitables, mais ils ont leur vertu pour

réponse. des marges de manœuvre prévues par le texte ? Je le répète, tout cadre implique une forme de rigidité. La condamner, c’est refuser le principe même d’un cadre. Nous assumons clairement le fait d’appeler à davantage de rigidité. Il faut bien sûr pouvoir ajuster le cadre à une situation exceptionnelle et imprévue. Lors de mes échanges avec des économistes, de hauts fonctionnaires et des professeurs de droit public, la question est apparue comme centrale. Le principal problème, c’est de décider qui peut déterminer, et par quel processus, qu’une situation doit

L’hypothèse est séduisante, mais elle pose un sérieux problème de légitimité démocratique. C’est pourquoi j’ai privilégié l’option d’un consensus politique, en retenant le mécanisme d’un vote à la majorité qualifiée. En 2020, au plus fort de la crise sanitaire, les budgets rectificatifs ont bien été adoptés en commission mixte paritaire. C’est donc bien par un consensus politique que la situation économique a été reconnue comme exceptionnelle et que des mesures exceptionnelles ont été prises pour y répondre. Il a également été dit que ce texte conduirait à renforcer le prétendu « gouvernement des juges », en conférant au Conseil constitutionnel la faculté de juger la conformité des lois de finances annuelles à la loi cadre. Mes chers collègues, le Conseil constitutionnel contrôle déjà la constitutionnalité des lois de finances Son rôle ne changerait donc pas. En revanche, son jugement serait éclairé par l’avis et l’expertise du Haut Conseil des finances publiques. C’est tout l’intérêt d’inscrire cet organisme dans la loi fondamentale.

Je n’ai pas la prétention d’apporter aujourd’hui un remède miracle contre le mal, non plus chronique, mais structurel, dont souffre la France. D’ailleurs, je m’en suis remise aux travaux déjà accomplis par ceux qui nous ont précédés. Ma proposition de loi constitutionnelle reprend ainsi la rédaction et l’architecture du projet de loi constitutionnelle de 2011, qui n’est pas allé à son terme. Ne rien faire ou faire comme si, un beau jour, bientôt, comme dans un conte de fées, la tendance lourde qui conduit à la dégradation de nos comptes publics allait soudainement s’inverser, par un heureux retournement de tendance, me semble irresponsable. Renoncer à un pilotage sur le long terme, c’est accepter d’être gouverné par le court terme, c’est préférer pour nos concitoyens la fragilité à la robustesse. Sans inverser le rapport entre annualité et pluriannualité, nous finirons toujours

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi constitutionnelle soulève un débat essentiel

l’absence de volonté de prendre des mesures concrètes afin de redresser nos finances publiques ; un échec juridique, ensuite, puisque cette proposition de loi constitutionnelle s’inspire grandement

Le troisième est de consacrer dans la Constitution le rôle du Haut Conseil des finances publiques tout en élargissant ses prérogatives. Le premier objectif,

toutefois, doit être manipulée avec la plus grande prudence, puisqu’il y a une différence de nature et de forme entre l’Union européenne et ses pays membres. L’Union européenne n’est pas un État souverain et ne joue pas un rôle majeur dans le fonctionnement des services publics.

J’ai conduit des auditions conjointement avec le rapporteur au fond, Stéphane Le Rudulier, et le rapport qu’il vient de faire reflète très bien les conclusions que j’ai moi même tirées de nos travaux. Depuis 1975, pas un seul budget n’a été voté à l’équilibre en France. La dégradation des comptes s’accélère, voire se banalise : depuis vingt ans, le déficit public n’a été inférieur à 3 % du PIB qu’à trois reprises. Chaque crise a fait franchir un nouveau palier à l’endettement public, qui ne parvient jamais à diminuer durablement 20 % à 40 % du PIB jusqu’au début des années 1990, 60 % après la récession de 1993, 80 % après la crise financière de 2009, il dépasse les 100 % depuis la crise de 2020. situation reflète un manque de volonté politique, surtout lorsque cette évolution perdure en sortie de crise ! En 2008, les lois de programmation des finances publiques ont été instituées afin d’infléchir cette tendance, mais les trajectoires qu’elles ont tracées n’ont pas été suivies. Face à l’échec des outils existants, je salue l’initiative de Vanina Paoli Gagin, qui nous amène à poser la question du redressement des finances publiques. La charge de la dette sera dans quelques années le premier poste de dépenses de l’État. Elle ampute ses marges de manœuvre et sa capacité à financer les transitions écologique, numérique ou démographique. Notre collègue nous propose d’instituer, pour la durée d’une législature, une loi portant cadre financier pluriannuel visant l’équilibre budgétaire et dont les dispositions s’imposeraient ensuite aux lois de finances annuelles, ainsi qu’aux lois de financement de la sécurité sociale. Sans reprendre toutes les analyses du rapporteur au fond, que je partage dans l’ensemble, je souligne que notre pays dispose déjà d’une Constitution financière, en quelque sorte : la loi organique relative aux lois de finances.

sur le respect par la loi de finances de la trajectoire des prélèvements obligatoires, par exemple, ou de la stratégie d’investissements publics fixées par la loi cadre, nous donnerions au juge de la Constitution le rôle d’un juge financier, voire d’un juge d’opportunité de la politique budgétaire. Ce n’est pas son rôle.

La procédure proposée ici aurait elle permis d’ouvrir des crédits en moins d’une semaine au mois de mars 2020 ? Je ne le pense pas. À l’inverse, une loi cadre votée en période d’euphorie pourrait acter des plafonds de dépenses excessifs.

Disons le : les règles juridiques ne peuvent pas remplacer la volonté politique. Ce débat nous permet de réaffirmer notre volonté de parvenir à infléchir la courbe du déficit et de l’endettement, mais la commission des finances ne vous propose pas d’adopter cette proposition de loi. La parole

Le Premier ministre a rappelé que la réduction du déficit public constitue une priorité absolue pour le Gouvernement. C’est l’objectif du projet de loi de finances pour 2025, que votre assemblée examinera bientôt. C’est dans ce contexte particulier que vous débattez de la proposition de loi constitutionnelle visant à accélérer le redressement des finances publiques. Ce texte ambitieux vise à modifier en profondeur les bases constitutionnelles de notre droit financier. Il prévoit de remplacer les actuelles lois de programmation des finances publiques par des lois portant cadre financier pluriannuel à caractère contraignant. Ces lois détermineraient pour une législature des plafonds de charge des administrations, des trajectoires de prélèvements obligatoires, des objectifs de solde public annuel et une stratégie d’investissement. Elles s’imposeraient aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, qui devraient, sous peine d’inconstitutionnalité, en respecter les orientations. Et ces lois cadres, dont la procédure d’adoption serait proche de celle des lois de finances actuelles, ne pourraient être modifiées qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres du Parlement réunis en Congrès. loi constitutionnelle interdit également l’adoption définitive d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale en l’absence de loi portant cadre financier pluriannuel. Elle renforce aussi les lois de finances en leur réservant le monopole des dispositions fiscales. Elle constitutionnalise les prérogatives du Haut Conseil des finances publiques et lui donne pour mission d’effectuer des prévisions économiques indépendantes. Elle impose un contrôle du Conseil constitutionnel sur tous les projets de loi financiers. Mme la

L’idée d’inscrire les choix budgétaires dans le temps long, et donc dans des normes d’application pluriannuelles, n’est pas nouvelle. Elle figure dans de nombreuses réflexions, auxquelles j’ai pu moi même participer au titre de précédentes fonctions, sur les moyens de concilier le principe d’annualité budgétaire avec la nécessaire prise en compte du temps long. Avant même l’apparition des lois de programmation, la pratique des débats d’orientation budgétaire permettait au Parlement de débattre des perspectives économiques et budgétaires des trois années suivantes et de fixer des objectifs d’évolution des dépenses. Nous avions voulu, avec Alain Lambert, conserver ce moment, utile à l’information du Parlement en matière budgétaire : il est désormais consacré par l’article 48 de la Lolf, qui prévoit la tenue d’un débat d’orientation des finances publiques en juillet devant les deux assemblées. Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) adopté en 1997 inscrit également les prévisions budgétaires dans un cadre pluriannuel, notamment au moyen du programme de stabilité transmis chaque année par le Gouvernement au Parlement et à la Commission européenne. l’outil de programmation pluriannuelle le plus abouti a vu le jour avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a introduit à l’article 34 de la Constitution les lois de programmation des finances publiques. Ces textes, en effet, définissent les orientations pluriannuelles des finances publiques, dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Cette formulation

Les lois de programmation définissent une trajectoire pluriannuelle, fixent des objectifs d’évolution du solde public et de la dette publique, en décrivant les perspectives relatives aux recettes et aux dépenses pour l’ensemble des administrations publiques, notamment des plafonds de crédits par mission du budget de l’État.

Cette loi organique a confié aux lois de programmation pluriannuelle des finances publiques le soin de fixer une trajectoire pluriannuelle. Elle a également créé le Haut Conseil des finances publiques, que j’ai eu l’honneur de présider, et qui veille au respect du principe de sincérité budgétaire consacré par l’article 32 de la Lolf.

publiquement le Parlement et le Gouvernement en cas d’écart avec la trajectoire fixée en loi d’orientation. Sur un plan juridique, donc, les lois de programmation des finances publiques sont aujourd’hui des instruments reconnus, à la fois utiles et nécessaires. utiles et nécessaires. Certes, ce sont aussi des instruments qui présentent certaines limites. En effet, par un saisissant paradoxe, les lois de programmation, qui ont vocation à traduire une vision de long terme, sont souvent celles qui sont le plus rapidement dépassées.

à la conduite des politiques publiques et à la bonne gouvernance des finances publiques ». C’est incontestable. Mais la prise en compte du temps long dans l’élaboration de la délibération démocratique, en particulier dans le domaine budgétaire, est particulièrement complexe. Elle doit en particulier être conciliée avec le principe de l’annualité budgétaire, ancré dans notre tradition politique et que je crois indispensable. Héritage de la révolution, ce principe permet à notre droit financier de se conformer aux exigences d’un régime démocratique représentatif. Le vote annuel des textes financiers garantit le respect des prérogatives du Parlement et l’effectivité de son contrôle. Et l’annualité permet d’ajuster les finances publiques à l’évolution de la croissance. Le Conseil constitutionnel a fait du principe d’annualité budgétaire un principe constitutionnel, qui découle des articles 34 et 47 de la Constitution. La nécessité de projeter la trajectoire financière dans un temps long, ou au moins sur le moyen terme, doit donc être conciliée avec ce principe. Cela pose inévitablement la question du rapport qui doit exister entre la loi de finances et la loi de programmation. En l’état du droit, le constituant a préféré faire des lois de programmation des instruments de pilotage et ne pas contraindre le Parlement dans le vote des lois de finances. Il faut dire que l’exercice est délicat. Les trajectoires fixées par les lois de programmation sont soumises par la suite à des contingences, notamment sociales, économiques, voire sanitaires récemment, qui ne peuvent être prises en compte au moment de leur élaboration, car elles ne sont pas toujours connues. connues. Ainsi, la trajectoire prévue par une loi de programmation est davantage une information sur la stratégie prévue à un moment donné par le pouvoir politique qu’une prévision de ce qui sera assurément et concrètement réalisé. Cette trajectoire constitue néanmoins un engagement qui lie politiquement le Gouvernement, en particulier aux yeux de nos partenaires européens. Faut il pour autant donner à ces instruments de programmation un caractère obligatoire et contraignant, comme le prévoit la présente proposition de loi constitutionnelle ? C’est ce qu’avait proposé le Président Nicolas Sarkozy dans le projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques déposé à l’Assemblée nationale le 16 mars 2011, que les deux assemblées ont voté dans les mêmes termes, mais qui n’a finalement pas été soumis au référendum ou au Parlement réuni en Congrès. Aujourd’hui, cette idée connaît un regain d’intérêt, alors que la situation de nos finances publiques est plus que préoccupante : la dette publique, vous l’avez rappelé, s’élève à plus de 3 000 milliards d’euros, soit plus de 110 % de notre PIB. Cette idée est séduisante en apparence, mais je ne peux pas y être favorable, et ce pour deux raisons. Premièrement, je pense qu’il ne faut pas minorer les inconvénients d’un système qui contraindrait juridiquement le Parlement et le Gouvernement dans leurs choix politiques. Ces dernières années l’ont démontré avec une vigueur particulière, sur le plan tant national qu’international : en dépit de toutes les prévisions et de tous les engagements, la politique financière reste tributaire des soubresauts de notre époque. Crises financières, pandémies, catastrophes naturelles ou encore guerres sont autant d’aléas que les politiques publiques doivent être capables d’appréhender. Le caractère non contraignant des lois de programmation des finances publiques offre une souplesse nécessaire au Parlement et au Gouvernement pour répondre rapidement à des situations d’urgence ou mettre en œuvre des politiques contracycliques, comme durant l’année 2020. Les solutions proposées dans cette proposition de loi constitutionnelle me paraissent affecter directement la capacité d’adaptation des pouvoirs publics. En définissant des indicateurs pour la durée de la législature, la loi cadre se révélerait fortement contraignante, notamment vis à vis de la politique budgétaire, qui reste utile en cas de ralentissement économique comme de récession. Par exemple, avec un plafond de charge fixé pour une législature, aucune réorientation ne serait possible sauf à convoquer le Congrès. La fixation de l’objectif de solde public pour une législature, alors que celui ci dépend pour beaucoup de la croissance, pourrait avoir un impact récessif. le nombre d’indicateurs susceptibles d’être modifiés au regard des aléas socio économiques souligne par lui même que le niveau constitutionnel n’est pas adapté pour un tel texte. De plus, il ne paraîtrait pas acceptable, en particulier pour nos concitoyens, que la représentation nationale se trouve privée de sa capacité de réaction parce qu’un texte programmatique aurait été voté des mois, voire des années plus tôt. La procédure d’adoption des lois cadres, et des textes financiers à leur suite, elle même rigide, ne permettrait pas de faire face à des situations d’urgence.

Enfin, la procédure de révision par les trois cinquièmes des membres du Parlement est particulièrement contraignante, sans que cela constitue une garantie de sérieux budgétaire. Je souscris pleinement, vous le savez, à l’objectif d’une plus grande maîtrise de nos finances publiques.

pour le pouvoir politique, qui doit garder la capacité de mener la politique budgétaire qu’il a déterminée et pouvoir réagir très rapidement si la situation l’impose. Les choix budgétaires demeurent avant tout des choix de nature politique, qui ne doivent pas être contraints par des outils juridiques

quelle qu’elle soit, restera toujours inefficace sans réelle volonté politique de rétablir nos comptes publics. La Lolf en est le meilleur exemple. De bons instruments juridiques ne peuvent suffire à faire baisser le niveau de déficit public et à assainir nos finances publiques : cela se saurait Il ne suffit malheureusement pas de changer les textes pour changer la réalité. Permettez moi de prendre l’exemple de deux de nos voisins les plus proches. L’Allemagne n’a pas attendu l’entrée en vigueur de l’interdiction constitutionnelle de voter un budget en déséquilibre, en 2016, pour redresser ses comptes publics.

pluriannualité dont nous avons besoin. Ce besoin, j’ai pu largement le rappeler dans le cadre de mes précédentes fonctions. En ce sens, je ne peux que saluer le vote de la loi organique du 28 décembre 2021, qui a précisé et modifié la Lolf et

Honnêtement, je ne le pense pas. Depuis sa création en 2014, il a déjà permis, par son influence et son expertise, de faire converger les prévisions du Gouvernement et celles du consensus économique, en particulier pour les prévisions de croissance, sans qu’il soit nécessaire de lui donner un cadre plus plus élevé dans la hiérarchie des normes. Son rôle pourrait toutefois, je le répète, être renforcé. Je suis persuadé que le redressement des comptes publics doit avant tout procéder de la volonté des acteurs politiques. Il nous appartient collectivement, membres du Gouvernement et du Parlement, de nous saisir de cette question cruciale. Les outils sont là. Il suffit de s’en saisir pour insuffler au sein des administrations une culture de la performance et de la responsabilisation des gestionnaires publics. Vous l’aurez compris, plutôt qu’à un nouveau big bang budgétaire, ou plus exactement de son cadre juridique, j’appelle bien plus volontiers à continuer les efforts qui ont été déployés dans le sillage de la Lolf et qui, pour beaucoup, restent à poursuivre, et à revenir à l’esprit

Permettez moi de dire que nous avons des marges de progrès considérables pour que cela corresponde à une réalité. À l’heure où les marges de manœuvre budgétaires semblent de plus en plus réduites, cet objectif me semble plus que jamais d’actualité. Nous devons nous efforcer de l’atteindre, bien sûr, sous le contrôle du Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai toujours été attaché au renforcement des prérogatives du Parlement en matière budgétaire et les fonctions que j’exerce aujourd’hui ne m’ont pas fait changer d’avis. Le rôle du Parlement dans le rétablissement de nos comptes publics me semble incontournable. Il possède à cet égard de puissants moyens d’information et de contrôle de l’action du Gouvernement, qui ne demandent qu’à être davantage utilisés.